d'entreprises, car elles ne disposent pas nécessairement des conseils juridiques dont bénéficient les grands groupes, la présidente de la CNIL a annoncé la publication prochaine d'une interface « clé en main », coproduite avec Bpifrance sous forme d'un « pack de conformité » au RGPD, destinée à ces acteurs. De manière générale, la mission d'information de la CNIL ne fait pas défaut, son trente-septième rapport annuel en témoigne. Il semble inapproprié aux sénateurs du groupe socialiste et républicain de commencer à compartimenter la mission générale d'information de la CNIL à ce stade. Il s'agit de la première mission de la CNIL et elle intéresse toutes les personnes concernées, qu'elles soient physiques ou morales, publiques ou privées. Il serait plus utile pour le Sénat, qui exerce une responsabilité particulière de représentation des collectivités territoriales, de mettre à profit la force de proposition de la CNIL pour suggérer au Gouvernement les mesures législatives et réglementaires d'adaptation de la protection des libertés à l'évolution des procédés et techniques informatiques, en prévoyant que cette mission particulière doive prendre en compte la situation des collectivités territoriales et celle des petites et moyennes entreprises.

En échange, les auteurs du présent amendement prévoient seulement que le rôle de veille législative de la CNIL pourrait lui permettre d'alerter le Gouvernement sur des mesures à prendre concernant les collectivités. Ce n'est pas du tout la même chose ! Nous sommes très attachés au rôle d'accompagnement de la CNIL auprès des petites collectivités et des petites structures. Je vous appelle donc à en rester au texte proposé par la commission.

une problématique également soulignée dans le rapport de la Cour des comptes de 2016 consacré à la « généralisation des services publics numériques ». Selon la Cour des comptes, les difficultés que rencontrent certains de nos concitoyens à manier les nouveaux outils numériques se doublent de difficultés liées à l'illettrisme classique. Or 90 % des contenus publiés sur internet prennent actuellement la forme de textes. Nous considérons qu'au même titre que d'autres publics vulnérables, tels que les mineurs, ces personnes devraient bénéficier d'une protection spécifique dans l'exercice de leur droit à la protection de leurs données personnelles.

sur la formation initiale et continue au numérique, par le numérique et avec le numérique, qui intègre toutes les générations, à commencer bien sûr par les enfants. Au cours des très nombreuses auditions que j'ai

ainsi libellé : La parole est à M. Alain Marc. Cet amendement vise à élargir le cadre des règlements types à la protection des données, par exemple au respect des droits en matière d'accessibilité, de finalité et de minimisation de la donnée. Cette rédaction permettra à la CNIL d'édicter des règlements de fond en matière de protection de la donnée et de respect de la vie privée. En novembre 2017, dans un avis sur la transposition de la directive européenne, elle avait fait la demande d'un élargissement du cadre des règlements types pour pouvoir élargir son champ d'action au-delà du seul sujet de la sécurité des systèmes. Ces nouvelles responsabilités consacrent son rôle de protecteur de la vie privée. Et Dieu sait si nous y sommes attachés au Sénat ! Outre l'accessibilité et la finalité des données, cet amendement vise à inscrire également dans le cadre des règlements types la question de la minimisation des données collectées. Il semble en effet opportun que la CNIL s'exprime et mette en oeuvre une règle de fond pour que la collecte et le traitement des données ne concernent que les données essentielles. Il s'agit d'une avancée importante pour le respect de la vie privée et des données personnelles. Quel est l'avis de la commission ? Cet

constitutionnel, car la délégation d'un pouvoir réglementaire aussi large à une autorité administrative risquerait d'être censurée au regard de l'article 21 de la Constitution. J'ajoute que la CNIL elle-même est satisfaite de la rédaction issue de l'Assemblée nationale et n'est pas demandeuse d'un nouvel élargissement de ses compétences sur ce point, ce qui est à mettre en rapport avec les arguments développés par Loïc Hervé tout à l'heure.

parole est à Mme Esther Benbassa. L'alinéa 11 de l'article 1prévoit que la CNIL établisse et publie des règlements types en vue d'assurer la sécurité des systèmes de traitement de données à caractère personnel, et de régir les traitements de données biométriques, génétiques et de santé. Dans ce cadre, elle peut prescrire des mesures techniques et organisationnelles supplémentaires pour le traitement des données biométriques, génétiques et de santé, conformément à l'article 9 du règlement européen, et des données relatives aux infractions pénales, conformément à l'article 10 du même règlement. L'alinéa 11 exclut ces mesures supplémentaires pour les traitements mis en oeuvre pour le compte de l'État agissant dans l'exercice de ses prérogatives de puissance publique. Nous ne partageons pas la philosophie de cette exception et considérons au contraire que, compte tenu de la nécessité d'encadrer strictement le traitement des données sensibles, il convient de la supprimer. La CNIL s'est d'ailleurs exprimée en ce sens dans sa délibération du 30 novembre 2017, regrettant notamment que les mesures techniques et organisationnelles supplémentaires qu'elle prescrirait pour le traitement de ces données « ne puissent concerner les traitements mis en oeuvre pour le compte de l'État, agissant dans l'exercice même des prérogatives

En effet, le présent article prévoit la possibilité de contraindre les collectivités territoriales, et non l'État, à prendre des mesures techniques et organisationnelles supplémentaires. Si la finalité de cette disposition est légitime, puisqu'elle vise à mieux protéger des données sensibles, en revanche il est incompréhensible

L'amendement n° 62 vise à étendre le champ d'application des garanties offertes par les règlements types de la CNIL aux traitements mis en oeuvre pour le compte de l'État en matière de génétique, de biométrique et de santé aux traitements de données. L'intention est louable, mais elle semble satisfaite par l'état du droit. En effet, si ces traitements sont hors du champ des règlements types de la CNIL, c'est qu'ils ne peuvent être créés que par un décret en Conseil d'État

à l'amendement n° 30, il vise à exempter les collectivités territoriales des garanties spécifiques que la CNIL peut imposer aux responsables de traitements de données biométriques, génétiques ou de santé. Cet amendement va beaucoup trop loin. Il s'agit de données particulièrement sensibles de nos concitoyens et, dans ce domaine, l'action de la CNIL est singulièrement la bienvenue. N'oublions pas que les règles de sécurité exigées par la CNIL concernant les données biométriques, génétiques et de santé sont aussi là pour protéger les élus locaux : en cas de problème, ils exposent leur responsabilité pénale. La commission demande le retrait

à l'État pour les traitements de données biométriques, génétiques et de santé. Comme Mme la rapporteur vient de l'indiquer, cela me semble difficile puisque les traitements de l'État sont soumis à une autorisation préalable, après avis de la CNIL.

Carrère. Si le projet de loi exclut effectivement l'État agissant dans l'exercice de ses prérogatives de puissance publique, c'est au motif qu'un régime contraignant existe à l'encontre de l'État. L'article 9 du projet de loi prévoit une formalité préalable particulière. Ces traitements, je le rappelle, sont autorisés par décret en Conseil d'État, pris après avis motivé et publié de la CNIL.

garde des sceaux. Le RGPD encourage la mise en place de mécanismes de certification pour faciliter la transparence et le respect du règlement, et permettre aux personnes concernées d'évaluer rapidement le niveau de protection des données offert par les produits et services proposés. Il s'agit donc d'une marge de manoeuvre pour la délivrance de l'agrément des organismes certificateurs. L'article 43 du RGPD prévoit en effet que cet agrément peut être délivré soit par l'autorité de contrôle- en France, il s'agit de la CNIL -, soit par l'organisme national d'accréditation-en France, le Comité français d'accréditation, le COFRAC -, soit par les deux. L'objectif du Gouvernement est de mettre en oeuvre cette marge de manoeuvre pour qu'au 25 mai 2018 la CNIL et le COFRAC soient en mesure de répondre à une forte demande prévisible d'agréments ou de certifications de manière directe. Or la rédaction actuelle du projet de loi, qui crée un bis à l'article 11 de la loi de 1978, ne répond pas totalement à cet objectif, car elle ne prévoit pas que le COFRAC puisse également agréer les certificateurs. C'est la raison pour laquelle nous avons déposé cet amendement, qui vise à introduire cette possibilité, étant précisé que la CNIL restera à l'initiative du choix de l'autorité chargée de cet agrément- soit elle-même ou Le Gouvernement propose par la même occasion de supprimer la dernière phrase de l'alinéa 13 selon laquelle la CNIL « peut établir des exigences supplémentaires en matière de normes d'accréditation ». Cette mention, qui est déjà prévue à l'article 43 du règlement de 2016, ne nous semble en effet pas nécessaire.

et de sécurité, et surtout le droit au « silence des puces », c'est-à-dire la possibilité de se déconnecter. Bien entendu, c'est au niveau européen qu'il importe d'avoir aussi une stratégie

le règlement ePrivacy est tout à fait nécessaire, mais il est loin d'être achevé ; on connaît aussi la lenteur des procédures. Il me semble que, pour tout mettre en cohérence par anticipation,

Parmi ceux que nous avons appelés les " naïfs " se trouvent d'abord les usagers, qui sont parfaitement conscients des capacités des acteurs du réseau à identifier, capter, manipuler leurs données et donc à analyser leur comportement, cerner leurs goûts et ainsi établir leur profil. » Car tel est bien l'objectif de l'objet connecté Mais, disent-ils, cela ne leur pose aucun problème, car " ils n'ont rien à cacher ni rien à se reprocher ". Précisons que ce syndrome du " rien-à-cacher-rien-à-me-reprocher " peut concerner aussi bien des familiers des moteurs de recherche et des réseaux sociaux que des personnes susceptibles de faire l'objet d'une prise de vue ou d'une géolocalisation, à leur insu ou non.

plus que rédactionnel. Il a pour objet de rendre effectif et non facultatif l'établissement de la liste des traitements susceptibles de créer un risque élevé

traitement susceptible, au regard de ses conclusions quant à l'analyse d'impact ou en raison de l'utilisation de nouvelles technologies, de présenter des risques élevés pour les droits et libertés des personnes concernées. Cet article prévoit que la CNIL peut établir une liste de ces traitements devant faire l'objet d'une consultation préalable. En prévoyant une simple faculté pour la CNIL d'établir cette liste de traitements non mis en oeuvre pour le compte de l'État, le projet de loi transpose strictement la directive.

pour tout traitement non mis en oeuvre par l'État dans le champ de la directive. En effet, si une autorisation de la CNIL est nécessaire pour créer tout traitement non mis en oeuvre par l'État dans le champ de la directive, il devient inutile de fixer une obligation de consultation préalable dans certains cas

Le présent amendement vise à étendre la possibilité de consulter la CNIL sur une proposition de loi ou sur toute disposition d'une proposition de loi relative à la protection des données personnelles, déjà prévue

comme toute autorité administrative indépendante, peut déjà répondre aux sollicitations ou solliciter directement le Parlement. Reste que, au moment où des propositions destinées à limiter les droits des parlementaires, à rendre le temps législatif expéditif ou à réduire l'influence

a pour objet de permettre aux présidents de groupe parlementaire de l'Assemblée nationale et du Sénat de saisir la CNIL sur toute proposition de loi ou sur toute disposition d'une proposition de loi relative à la protection ou au traitement des données à caractère personnel.

L'opposition n'est pas à la mode ; on le constate à chaque annonce relative à la réforme des institutions, et la restriction du droit d'amendement en est un exemple flagrant. Mais l'opposition existe

toute autre autorité ou institution intéressée par l'accomplissement de ses missions. Il s'agit de favoriser le dialogue entre les différentes autorités ou institutions compétentes sur les problèmes numériques. Quel est l'avis de la commission ? La faculté de saisine d'une autorité indépendante par une autre est consacrée et généralisée par leur statut général, voté sur l'initiative de notre assemblée. L'amendement étant sans objet, j'en demande le retrait.

Robert. Cet amendement ouvre un débat et soulève un enjeu démocratique relatif au statut et au rôle que pourraient être amenés à jouer les futurs délégués à la protection des données. En un sens, le délégué à la protection des données- ou DPO, pour sera la clé de voûte de l'application du règlement : à la fois conseiller du responsable, mais aussi du sous-traitant mettant en oeuvre le traitement, garant du respect des obligations leur incombant et point de contact de l'autorité de contrôle ainsi que des citoyens s'enquérant d'une information, il occupera une occupera une position stratégique et aura une vision synoptique. Il sera donc en mesure de déceler d'éventuels manquements ou violations liés à la protection des données personnelles, sous réserve que lui soient garanties des conditions idoines à l'exercice de ses missions, notamment, bien sûr, en termes d'indépendance. Dans les cas les plus graves- songeons aux

où les atteintes aux droits sont à la fois massives par leur ampleur et considérables par leur nature, il s'avère essentiel de permettre au délégué de jouer pleinement son rôle de vigie, voire de révélateur de pratiques contraires aux droits fondamentaux. C'est pourquoi les auteurs de cet amendement proposent que, lorsque le délégué à la protection des données signale, de manière désintéressée et de bonne foi, des violations graves, manifestes et répétées des droits et libertés mentionnés à l'article 1 de la loi du 6 janvier 1978, il puisse bénéficier du statut de lanceur d'alerte créé par la loi Sapin II.

que « le responsable du traitement et le sous-traitant veillent à ce que le délégué à la protection des données ne reçoive aucune instruction en ce qui concerne l'exercice de ses missions ».

Le présent amendement vise à introduire plus de souplesse dans l'organisation interne des travaux de la CNIL. Son adoption permettrait à la formation plénière de la commission de déléguer au président ou au vice-président délégué certaines décisions touchant aux nouvelles obligations de notification des violations de données. Conformément à l'article 34 du RGPD, la CNIL devra recevoir ces notifications et examiner si la violation est susceptible d'engendrer un risque élevé, afin soit d'exiger du responsable de traitement de communiquer cette violation aux personnes concernées, soit de décider que cette communication n'est pas nécessaire. Les services de la CNIL ont mis en avant auprès de votre rapporteur les chiffres des Pays-Bas, où cette obligation de notification existe déjà en droit positif : 6 500 notifications par an, dans un pays bien plus petit que la France. Il convient d'aider la CNIL à ménager ses moyens en lui offrant cette agilité organisationnelle.

madame la ministre, mes chers collègues, les travaux antérieurs du groupe du RDSE sur les autorités administratives indépendantes et leur fonctionnement. Le projet de loi introduit de nouvelles dispositions visant à encadrer le rôle du commissaire du Gouvernement siégeant auprès de la CNIL et désigné par le Premier ministre. Dans la même logique, nous considérons que, pour respecter la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme et la théorie des apparences, il serait utile de le renommer, comme on l'a fait au sein de la juridiction administrative. administrative. Les personnes visées par les sanctions prononcées par la CNIL doivent avoir la certitude que ces sanctions ont été prononcées en toute indépendance, sans que le commissaire du Gouvernement donne l'impression d'avoir pesé dans la décision de sanction.

l'article 90 du RGPD. Cet article autorise l'adoption de règles spécifiques, afin de définir les pouvoirs des autorités de contrôle à l'égard des responsables du traitement ou des sous-traitants, qui sont soumis à une obligation de secret professionnel ou à d'autres obligations de secret équivalentes, lorsque cela est nécessaire et proportionné, et ce pour concilier le droit à la protection des données à caractère personnel et l'obligation de secret. Notre amendement vise à prendre en compte le cas des données couvertes par le secret professionnel, lorsque ces dernières sont stockées et traitées par un fournisseur de service dans le cadre d'un contrat de, le problème étant que les données ne sont pas stockées dans les serveurs eux-mêmes objets du contrôle.

ou de traitements, ou de la gestion de service de santé, réalisée dans le cadre de ce contrôle. Toutefois, il prévoit que la communication de ces données médicales ne pourra plus être requise obligatoirement par un médecin, comme le prévoit le droit en vigueur, mais sous son autorité et en sa présence. Cet assouplissement de la procédure de requête représente un recul par rapport au droit existant. Compte tenu de la nature même des données médicales qui leur confère une sensibilité particulière, il convient de laisser le médecin jouer le premier rôle et de s'assurer de son autonomie de jugement.

de la recherche médicale, des diagnostics médicaux, de l'administration de soins ou de traitements, ou de la gestion de service de santé ne peut se faire qu'après information préalable du patient. Il vise ainsi à respecter le principe de transparence à l'égard des personnes concernées, lequel régit l'ensemble du règlement 2016/679.

Le texte du projet de loi est légèrement moins strict : il prévoit dans un tel cas que la communication des données ne pourra désormais se faire que « sous l'autorité et en présence d'un médecin ». Comme le précise l'avis du Conseil d'État, qui est à l'origine de la rédaction retenue, l'agent menant le contrôle sera placé sous la responsabilité fonctionnelle du médecin, qui ne réalisera pas nécessairement lui-même les opérations informatiques, mais adressera toutes les instructions nécessaires à l'agent pour que ne soit pas violé le secret médical Les garanties déjà prévues dans le texte de la commission me semblent importantes, car elles concilient à la fois l'exigence de préservation du secret médical et la nécessaire efficacité opérationnelle des contrôles de la CNIL.

protecteur pour la personne concernée, laquelle peut d'ailleurs être à l'origine du contrôle, maintiendrait les difficultés procédurales relevées par la CNIL, alors même que l'accroissement de ses missions nécessite- nous l'avons dit à plusieurs reprises -d'en optimiser les ressources. C'est la raison pour laquelle le Gouvernement a souhaité modifier le régime procédural en prévoyant désormais que la communication des données médicales individuelles ne pourra se faire que sous l'autorité et en présence d'un médecin. Cette rédaction issue de l'examen du projet de loi au Conseil d'État signifie que l'agent menant le contrôle sera placé sous la responsabilité fonctionnelle du médecin,

dans le cadre du déroulement des contrôles, à la fois dans le temps et dans la forme, ou bien dans certains cas comme, par exemple, lorsque la personne est dans l'incapacité au regard de son état de santé de recevoir l'information.

: La parole est à Mme la garde des sceaux. Cet amendement vise à réintroduire la possibilité pour les membres et les agents de la CNIL de faire appel à des experts dans le cadre de leurs opérations de contrôle. Il s'agit de rétablir une possibilité déjà prévue par les dispositions de l'article 44 de la loi de 1978

pour contrôler les opérateurs de jeux en ligne. L'adoption du présent amendement offrirait l'occasion d'élargir le recours aux experts en supprimant la condition imposant leur désignation préalable par une autorité.

et notamment des fichiers qu'ils produisent, qu'il s'agisse de l'usage des techniques de renseignement ou de leur résultat en termes de données collectées et traitées, répond à une exigence légitime pour tous ceux qui sont attachés au respect des droits de l'homme. Bien que ces fichiers ne soient soumis ni au RGPD ni à la directive que le présent projet de loi entend transposer, les modalités de leur contrôle présentent un lien direct avec le texte que nous examinons, dès lors que l'article 4 du projet de loi modifie l'article 44 de la loi de 1978 dont le IV prévoit, en l'état actuel du droit, que les pouvoirs de contrôle général des fichiers reconnus à la CNIL ne s'appliquent pas à certains traitements intéressant la sûreté de l'État. En conséquence, pour un certain nombre de fichiers considérés comme stratégiques, la possibilité pour la CNIL d'opérer un contrôle sur pièce et sur place, plein et entier, est exclue à ce jour. Certes, il s'agit de données sensibles au sens où elles intéressent directement la sûreté de l'État, la défense et la sécurité publique. D'ailleurs, elles bénéficient déjà à ce titre d'un régime largement dérogatoire et tout à fait justifié. Par ailleurs, des garde-fous ont été institués par la loi du 24 juillet 2015 relative au renseignement. La Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement, la CNCTR, autorité administrative indépendante, est appelée à émettre un avis préalablement à la mise en oeuvre d'une technique de renseignement susceptible d'alimenter ces fichiers. Celle-ci procède également à des contrôles. Toutefois, la CNCTR ne s'occupe que des techniques par le biais desquelles les fichiers sont alimentés et n'exerce son contrôle qu'au regard du cadre juridique rigoureux élaboré par le législateur dans le cadre de la loi du 24 juillet 2015. Telle est sa mission et c'est déjà beaucoup ! En revanche, la CNCTR n'est pas compétente pour juger du respect de la protection des données personnelles dans le champ de la loi du 6 janvier 1978. Actuellement, il existe bien vide juridique, dans la mesure où aucun contrôle de ces fichiers, qui permettrait de garantir leur mise en oeuvre dans le respect de la protection des données personnelles et des textes applicables en la matière, auxquels ils sont pourtant soumis, n'est prévu. L'adoption de cet amendement contribuera à accroître la confiance des citoyens dans l'action des services de renseignement, à diffuser et conforter la culture du renseignement que nous souhaitons promouvoir avec force et,, à renforcer la sécurité de tous dans le respect des libertés publiques.

ce contrôle ne ferait qu'affaiblir nos services de renseignement et risquerait de dissuader nos partenaires de nous transmettre des informations. J'ajoute

les fichiers de renseignement constituent un sous-ensemble des fichiers dits « de souveraineté », qui intéressent la sûreté de l'État, la défense et la sécurité publique, et qui sont mentionnés à l'article 26 de la loi Informatique et libertés. De par la nature même de ces fichiers et les finalités qu'ils servent, certains droits ne sont pas reconnus aux personnes concernées. Le droit d'accès aux données contenues dans ces traitements est ainsi exclu. Néanmoins, toute personne qui s'interroge sur la présence dans ces fichiers de données la concernant peut s'adresser à la CNIL, qui procédera aux vérifications en son lieu et place. C'est ce que l'on appelle le « droit d'accès indirect ». Les principales caractéristiques de ces fichiers de renseignement-

pour des raisons évidentes de confidentialité, et afin de ne pas mettre en cause leur finalité même, la plupart de ces décrets sont dispensés de publication, comme l'autorise l'article 26 de la loi Informatique et libertés. Le décret du 15 mai 2007 liste les quatorze fichiers concernés par ces dispositions. La possibilité pour la CNIL d'opérer un contrôle sur pièce et sur place, plein et entier, n'est exclue que pour huit de ces quatorze fichiers : il ne s'agit donc que des fichiers de renseignement les plus sensibles et pour lesquels la possibilité d'obtenir copie de tout document ou information et d'examiner l'architecture des outils techniques est exclue, au risque de mettre gravement en cause les modalités d'action des services de renseignement. Au demeurant, l'accès à ces fichiers au sein des services de renseignement est étroitement encadré par des habilitations précises le dispositif de l'amendement pourrait mettre en cause les modalités d'action des services de renseignement, mais aussi le lien de confiance entre nos services et les services étrangers partenaires. Ce n'est qu'avec l'accord exprès d'un partenaire que l'on peut mettre des informations qu'il a partagées à la disposition d'un tiers. Les huit fichiers dont je viens de parler relèvent de la DGSE, pour deux d'entre eux, de la DGSI et de la Direction du renseignement militaire,

Si, les concernant, la CNIL ne peut pas effectuer un contrôle plein et entier de droit commun, il n'en demeure pas moins que ces fichiers font déjà l'objet d'une pluralité de contrôles.

du respect des conditions posées par l'autorisation. Ce contrôle est réalisé pour chaque service deux à trois fois par mois de manière très approfondie. Il se double d'ailleurs d'un dialogue très exigeant entre la CNCTR

il ne faut pas l'oublier, la création de ce fichier est subordonnée en amont à un examen préalable de la CNIL, puis à celui du Conseil d'État qui, pour autoriser la création par décret de ce traitement, s'assure de la légalité de ses principales caractéristiques, type de données recueillies, leurs modalités de conservation et les possibilités de croisement. Une fois ce fichier créé, et dans le cadre du droit d'accès indirect que j'ai précédemment évoqué, la CNIL se rend trois à quatre fois par an dans chacun des services de renseignement afin de vérifier, au bénéfice des personnes qui la saisissent, que les données détenues le cas échéant par ces services sont nécessaires et respectent les caractéristiques initialement définies dans le texte réglementaire sur lequel la CNIL a donné son avis. Ce contrôle fait par la suite l'objet de nombreux échanges entre le service de renseignement concerné et la CNIL afin, le cas échéant, de procéder à la rectification ou à l'effacement des données qui ne seraient pas pertinentes. Enfin, une personne qui pense être connue d'un service de renseignement peut, sans autre condition préalable que le soupçon qui l'habite, saisir une formation spécialisée du Conseil d'État habilitée au secret de la défense nationale, afin d'obtenir l'effacement des données la concernant si celles-ci sont irrégulièrement détenues par les services de renseignement. À l'occasion de ce recours, la CNIL intervient systématiquement et produit les éléments qu'elle a recueillis lors de l'exercice du droit d'accès indirect. Il me semble que cette pluralité de contrôles répond à une logique propre, qui a été définie à l'occasion de l'adoption de la loi de 2015 relative au renseignement. la CNCTR est compétente pour contrôler le recueil des données brutes de renseignement, c'est-à-dire celles qui seront saisies à l'occasion de l'utilisation d'une technique de renseignement. La CNIL, quant à elle, est compétente pour contrôler les conditions dans lesquelles les données recueillies sont conservées et, surtout, les conditions dans lesquelles celles-ci sont exploitées dans un fichier. Cette ligne de partage voulue par le législateur est essentielle, puisque les activités des services de renseignement ne sont pas les mêmes. Si les membres et les agents de la CNCTR, ceux de la CNIL, sont habilités au secret de la défense nationale, le principe du cloisonnement en matière de renseignement, qui s'applique au fonctionnement quotidien des services comme aux relations avec nos partenaires étrangers,

Carrère. L'article 4 du projet de loi précise les conditions dans lesquelles les agents de la CNIL sont autorisés à contrôler les traitements de données réalisés par les juridictions, sans lien avec leur fonction juridictionnelle. S'agissant des contrôles des traitements de données médicales stockées par les médecins, qui sont mentionnés au même article du projet de loi, le texte introduit une garantie supplémentaire, à savoir la présence d'un médecin lors des contrôles ainsi conduits par la CNIL, afin de préserver le secret médical. Nous considérons que le secret de l'instruction devrait également être protégé dans des conditions comparables. C'est pourquoi nous proposons, par mimétisme avec le dispositif que je viens d'évoquer, que les contrôles des agents de la CNIL se fassent en présence et sous l'autorité d'un magistrat. Cela permettrait de s'assurer que ces contrôles ne concernent que le traitement des données, sans lien avec la fonction juridictionnelle.

dispositif de l'amendement est un peu ambiguë. Il n'est pas précisé si le magistrat ainsi chargé du contrôle sera membre de la CNIL ou bien de la juridiction concernée par le contrôle. Dans le premier cas, cela pourrait occasionner des difficultés opérationnelles,

d'abord, un avertissement en cas de simple risque de manquement, puis une mise en demeure en cas de manquement encore susceptible de faire l'objet d'une mise en conformité et, enfin, une procédure de sanction. Après avoir consulté la CNIL, qui souhaitait conserver une marge d'appréciation et préserver les dispositifs de coopération avec ses homologues, nous sommes parvenus, avec cet amendement de compromis, à une rédaction respectueuse de la liberté d'action de l'autorité, mais plus pédagogique que celle du texte initial.

Contrairement aux grands groupes, l'adaptation à ces nouvelles normes dans les petites structures dépourvues de service juridique interne sera probablement plus laborieuse, sans pour autant que cette phase transitoire représente un risque d'utilisation illicite des données personnelles supérieur au risque actuel. du 2 de l'article 83 du RGPD prévoit spécifiquement de tenir compte, pour le prononcé de l'amende, du fait que la violation a été commise délibérément ou par négligence. délibérément ou par négligence. De ce point de vue, l'introduction d'une présomption de négligence en faveur des petites et moyennes entreprises est conforme à l'esprit de l'article que d'adopter représente certes une atténuation du principe d'égalité, mais nous paraît justifiée au regard de la situation particulière dans laquelle se trouvent les petites entreprises dépourvues de services informatique ou juridique suffisants.

qui prévoit que le produit des amendes et des astreintes prononcées par la CNIL est destiné à financer l'assistance apportée par l'État aux responsables de traitement et à leurs sous-traitants, afin que ceux-ci se conforment aux obligations en vigueur en matière de protection des données.

que dans le cadre des procédures prévues en son article 16. Tout à fait ! Selon cet article, certaines recettes peuvent être directement affectées à certaines dépenses, et ces affectations prennent la forme de budgets annexes. Or, en l'espèce, ces modalités d'affectation ne semblent pas avoir été respectées.

relève en premier lieu de la CNIL. L'article 57 du RGPD donne en effet à l'autorité de contrôle, en l'occurrence la CNIL, la mission d'encourager « la sensibilisation des responsables du traitement et des sous-traitants en ce qui concerne les obligations qui leur incombent en vertu du présent règlement ».

doit résulter d'une disposition de loi de finances. À l'heure actuelle, le produit de l'ensemble des amendes prononcées par les autorités administratives

Cet amendement vise uniquement à harmoniser le niveau des amendes. L'article 83 du RGPD punit d'une amende pouvant s'élever jusqu'à 20 millions d'euros, ou 4 % du chiffre d'affaires annuel mondial, le non-respect des pouvoirs d'enquête de l'autorité de contrôle, c'est-à-dire de la CNIL.

Par ailleurs, les contraventions prévues dans les articles réglementaires du code pénal aux articles R. 625-10 à R. 625-13, et qui relèvent d'un décret en Conseil d'État, visent des faits classés par le RGPD parmi les manquements les plus graves. Ces faits devraient donc être requalifiés en délits,

applicables en cas de non-respect des règles relatives à la protection des données personnelles. Il nous semble néanmoins difficile de souscrire aux qualifications et peines proposées, qui apparaissent manifestement excessives.

que nous nous imposerons. La création d'une coopération entre autorités de contrôle n'aura pas d'effet positif sur la protection des données personnelles des citoyens européens si certains États membres adoptent des stratégies non coopératives. Il est à prévoir que la mise en oeuvre de cette coopération puisse, dans les premiers temps de l'application, donner lieu à certains flottements, tant le mécanisme est innovant. Cette réciprocité est d'autant plus nécessaire que, jusqu'à présent, le législateur français s'est appliqué à assurer un niveau très élevé de protection des données personnelles. est l'avis de la commission ? La commission demande le retrait de cet amendement, contraire au règlement général européen. Celui-ci, d'application directe, détermine de façon complète les obligations de coopération et d'assistance mutuelle que se doivent les différentes autorités européennes.

à une demande d'assistance, sauf si « satisfaire à la demande constituerait une violation du présent règlement ou du droit de l'Union ou du droit de l'État membre auquel l'autorité de contrôle qui a reçu la demande est soumise

à M. Jérôme Durain. Le RGPD renforce la coopération européenne en matière de protection des données personnelles. Il instaure un système d'action cohérente et d'assistance mutuelle entre les différentes autorités compétentes. Dans ce cadre, la CNIL pourra être amenée à réaliser des opérations conjointes avec les autorités de contrôle des autres États membres. Lorsqu'une opération de contrôle conjointe se déroule sur le territoire français, les membres et agents de la CNIL sont présents aux côtés des membres et agents des autres autorités de contrôle participant à l'opération. Le droit national s'impose. Il ressort en effet de la négociation du RGPD le souci des États membres de veiller au respect de la souveraineté nationale. À cet égard, le règlement prévoit une marge de manoeuvre laissée aux États membres concernant les pouvoirs d'enquête confiés aux membres et agents associés aux opérations conjointes. En conséquence, lorsque le président de la CNIL habilite les membres et agents de ces autorités à participer à des opérations se déroulant sur le territoire national, il convient de préciser que ces derniers exercent sous son autorité, mais également sous son contrôle, tout ou partie des pouvoirs de vérification et d'enquête dont disposent les agents de la CNIL.

L'article 5 du projet de loi, dans sa rédaction actuelle, est conforme au règlement de l'Union européenne et il n'est pas nécessaire, de mon point de vue, d'effectuer l'ajout proposé, dès lors que les autres États membres n'adopteraient pas une rédaction similaire.

Le délégué à la protection des données est chargé de mettre en oeuvre la conformité au règlement général sur la protection des données au sein de l'organisme qui l'a désigné, et ce pour l'ensemble des traitements auxquels cet organisme La désignation d'un délégué est obligatoire pour les autorités ou les organismes publics. Elle s'effectue sur la base de ses qualités professionnelles et, en particulier, de ses connaissances spécialisées du droit et des pratiques en matière de protection des données, et de sa capacité à accomplir ses missions. Du fait de ces attributions sensibles, il semble cohérent que le mouvement déontologique à l'oeuvre dans l'ensemble de la sphère publique s'applique également à la fonction de DPO. La particularité de son office plaide également pour des dispositions déontologiques spécifiques, que la CNIL serait le plus à même d'identifier. Un tel document, associé aux chartes existant déjà dans le secteur privé, pourrait en outre contribuer à mieux définir les bonnes pratiques pour l'ensemble des DPO.

personnel révélant la prétendue origine raciale ou l'origine ethnique, les opinions politiques, les convictions religieuses ou philosophiques

Marc. Cet amendement tend à protéger les jeunes élèves en instituant une interdiction de traitement des données à caractère personnel collectées dans le cadre de l'utilisation de services numériques au sein de l'éducation nationale. Il vise à inscrire dans le droit une obligation souvent présente dans les conditions générales d'utilisation des services numériques de l'éducation nationale. La protection de la vie privée et des données personnelles des élèves du premier et du second cycles est essentielle et ne peut être négligée. Il faut donc instituer une véritable protection pour ces publics fragiles, souvent imprudents, sur les supports numériques, avec leurs données personnelles. Quel est l'avis de la commission ? Cet amendement aborde un point important. Néanmoins, sa rédaction est beaucoup trop large et l'interdiction proposée risque de paralyser l'activité des établissements, où la gestion des élèves et des notes

à savoir garantir aux élèves et à leurs familles la protection des données personnelles collectées dans le cadre scolaire. Il s'agit d'ailleurs d'une priorité de la politique conduite par le ministère de l'éducation nationale en matière de développement des outils numériques. Je rappelle que le ministère, je l'indiquais dans mon propos introductif, a mis en oeuvre un traitement de données personnelles dénommé « Gestionnaire d'accès aux ressources », », dont l'objet est de rationaliser la communication des données aux fournisseurs de ressources ou de services. Cet outil permet donc, en vue de respecter le principe de minimisation des données, de ne transmettre aux fournisseurs de ressources ou de services que des données strictement nécessaires aux accès des élèves et des enseignants à ces ressources. L'amendement proposé porte sur l'ensemble des données collectées dans le cadre de l'utilisation de services numériques au sein de l'éducation nationale. Il concerne donc potentiellement tous les services numériques utilisés dans les établissements scolaires

On a parlé des petites communes, des petites associations, des petites entreprises, mais, là, on parle d'un grand employeur public, l'un des plus grands du monde après l'armée chinoise : l'éducation nationale.

de corriger certaines contradictions entre le projet de loi et le règlement. L'article 9 du RGPD manque de précision en n'interdisant pas explicitement les traitements qui, recoupant des données non sensibles que la personne concernée a publiées, visent à reconstituer des données sensibles, qui, elles, n'ont jamais été publiées par la personne. De même, cet article n'autorise le traitement de données sensibles que pour certaines finalités dont il dresse la liste exhaustive. Or l'article 8 de la loi de 1978, tel que modifié par le projet de loi, autoriserait les traitements de données sensibles poursuivant n'importe quelle finalité, pour la simple raison qu'une mesure technique serait appliquée : l'anonymisation à bref délai. Cela n'est pas autorisé par le RGPD : cette autorisation doit être limitée à des finalités précises. Cette contradiction doit par conséquent être supprimée. cette mesure d'anonymisation à bref délai n'est pas sans intérêt. En effet, l'article 9 du RGPD prévoit que, s'agissant de certaines finalités, le traitement de données sensibles n'est licite qu'en présence de « mesures appropriées et spécifiques pour la sauvegarde des droits fondamentaux et des intérêts de la personne concernée Pour certaines de ces finalités, la loi de 1978 prévoit effectivement des garanties qui pourraient correspondre à ces « mesures appropriées ». Néanmoins, s'agissant d'autres finalités- celles visées au, et du 2 de l'article 9 du règlement -, la loi n'en prévoit aucune. Ainsi, dans ce cas précis, la mesure d'anonymisation à bref délai pourrait être une des « mesures appropriées » autorisant la poursuite de ces finalités.

en interdisant de manière explicite les traitements qui visent à reconstituer des données sensibles qui n'ont jamais été publiées par la personne. D'autre part, il tend à corriger une contradiction entre le présent projet de loi et le règlement européen. En effet, l'article 9 du règlement général sur la protection des données n'autorise le traitement de données sensibles que pour certaines finalités dont il dresse une liste exhaustive. de 1978 tel que modifié par le projet de loi, reviendrait à autoriser en cas d'application d'une mesure technique telle l'anonymisation à bref délai les traitements de données sensibles poursuivant n'importe quelle finalité. Nous considérons que cela est contraire au RGPD : cette autorisation doit être limitée à des finalités précises.

qui, comme vous le savez, est d'application immédiate et totale, sauf s'il est prévu une marge de manoeuvre, ce qui ne me semble pas être le cas en l'espèce. Par ailleurs, ainsi que cela a été indiqué en réponse à l'amendement n° 137, la précision est inutile dès lors qu'est interdit tout traitement qui révèle une donnée sensible au sens de l'article 9 du RGPD. D'autre part, la dérogation au traitement des données sensibles, si ces traitements font l'objet à bref délai d'un procédé d'anonymisation, est, dans la rédaction du projet de loi, compatible avec le RGPD. Cette disposition, cela vient d'être souligné, est prévue actuellement par l'article 8 de la loi de 1978, je rappelle que ce procédé d'anonymisation devra avoir été préalablement reconnu conforme à la présente loi par la CNIL. Celle-ci sera vigilante sur la compatibilité de ce processus avec le RGPD. En outre, cette anonymisation à bref délai sera également utile pour les traitements qui ne relèvent ni du règlement ni de la directive. Il ne semble donc pas pertinent de restreindre le champ de l'anonymisation, comme cela est proposé. La parole est

Jourda. Cet amendement vise à autoriser les établissements financiers à utiliser les données biométriques qui leur sont nécessaires pour identifier leurs clients dans le cadre de l'obligation de vigilance qui leur est faite par l'ordonnance du 1 décembre 2016.

permettre aux établissements financiers d'utiliser des bases de données biométriques pour les aider à remplir les obligations de vigilance qui leur sont imposées par le code monétaire et financier. Ces obligations consistent essentiellement en une

En l'état du droit, il me semble que rien n'est prévu spécifiquement pour les autoriser à mettre en oeuvre des traitements de données biométriques. Autoriser de tels traitements demanderait, surtout pour des acteurs privés, de robustes garanties que cet amendement ne propose pas. Nous n'avons pas assez de recul sur la portée sur la portée d'une telle dérogation pour l'autoriser sans mener une réflexion plus approfondie. La CNIL, qui a été consultée, souligne la complexité du sujet et recommande la prudence. Quel est l'avis du Gouvernement ? est défavorable. Cet amendement me semble en effet excessif dans sa portée. Madame la sénatrice, vous souhaitez que les établissements financiers bénéficient de droits, mais sans être soumis à la moindre formalité. Ces droits, de par leur ampleur et en raison de leurs contours indéfinis, ne sont accordés ni à l'État par le RGPD ni par la directive aux autorités qui sont directement chargées de la lutte contre le blanchiment d'argent et le terrorisme. d'une telle mesure dans l'article 8 de la loi de 1978 accorderait une dérogation générale, non seulement pour les données biométriques, mais aussi pour toutes les données sensibles au sens du RGPD.

lorsqu'elles ne peuvent s'appuyer sur le consentement des personnes concernées, sont majoritairement soumises à l'autorisation préalable de la CNIL, en application des dispositions du IV de l'article 8 et de celles de l'article 25 de la loi du 6 janvier 1978. Dans sa rédaction actuelle, le projet de loi supprime l'article 25, ce qui a pour conséquence de soumettre ces traitements à un dispositif d'autorisation par décret en Conseil d'État, pris après avis motivé et publié de la CNIL. Cette procédure nous semble particulièrement problématique, surtout pour les chercheurs, et constitue une véritable entrave à la recherche publique. Nous proposons donc, à l'instar du Gouvernement, d'instaurer une exception pour cette dernière dans la mesure où les traitements à finalité de recherche publique

dans le champ des exceptions à l'interdiction de traitement des données sensibles hors consentement de la personne concernée. À l'heure actuelle, seuls les traitements statistiques réalisés par l'Institut national de la statistique et des études économiques ou l'un des services statistiques ministériels les traitements qui sont nécessaires à la recherche, aux études et aux évaluations dans le domaine de la santé sont couverts par les exceptions prévues au 7° et 8° du II de l'article 8. Les autres traitements de la recherche publique sont soumis à une autorisation préalable de la CNIL. Tel est le cas en particulier d'un grand nombre d'études qui sont menées dans le champ de la sociologie ou de la démographie- je pense notamment aux enquêtes portant sur les migrants ou bien encore sur les violences faites aux femmes. L'abrogation de l'article 25 de la loi de 1978 par le projet de loi dans la logique d'allégement des formalités préalables a pour conséquence de soumettre ces traitements à un dispositif d'autorisation par décret en Conseil d'État, après un avis motivé et publié de la CNIL. Une telle formalité apparaît sans doute beaucoup trop lourde et très rigide s'agissant de ce type de traitements. Il est donc proposé d'inscrire au titre des exceptions énumérées au II de l'article 8 un alinéa supplémentaire relatif à la recherche publique prise au sens de l'article L. 112-1 du code de la recherche. Une telle dérogation est permise par le RGPD, qui la prévoit pour les traitements d'intérêt public importants ou pour des fins de recherche scientifique. En contrepartie de la suppression de l'article 25, il est prévu que la CNIL soit consultée au préalable et que son avis soit motivé et publié. Quel est l'avis de la commission ? Avis favorable.

la loi Informatique et libertés n'auront pas vocation à régir les traitements soumis au règlement, qui est d'application directe et fixe lui-même son champ d'application territorial.

lorsque celle-ci sera appliquée de façon complémentaire au nouveau règlement européen, dans le but de le rapprocher tout à la fois du critère d'application du règlement européen lui-même et du critère d'application de la même loi de 1978 lorsqu'elle est appliquée seule, indépendamment du règlement. Il résulte en effet de l'article 8 du projet de loi en sa rédaction actuelle un degré de complexité qui paraît incompatible avec les exigences de lisibilité et de bonne application de la loi, exigences d'autant plus impérieuses lorsque celle-ci vise à protéger les droits et libertés des personnes physiques. L'article 8 prévoit, dans la version du projet de loi adoptée par l'Assemblée nationale, un champ d'application de la loi de 1978 centré sur la résidence de la personne dont les données sont traitées, dans les cas où cette loi vient préciser les dispositions du règlement en application des marges de manoeuvre laissées aux États membres de l'Union européenne par ce dernier. le règlement européen se réfère systématiquement en principe au critère d'établissement non pas de la personne concernée, mais du responsable du traitement. Par exception, dans certains cas limités, le règlement européen sera par ailleurs applicable lorsque ce responsable de traitement sera établi hors de l'Union européenne, sous réserve que la personne concernée soit localisée en France, la notion de localisation se distinguant de celle de résidence. Cet éclatement des critères risque d'entraîner une confusion importante dans l'application territoriale de la loi de 1978, notamment de la part des entreprises et organismes publics responsables de traitements, qui ne seront pas en mesure d'identifier facilement les règles de droit qui leur sont applicables. Par ailleurs, le choix d'un critère de résidence de la personne concernée a pour effet d'imposer systématiquement la collecte de l'adresse de cette personne, même dans les cas où cette donnée n'est pas nécessaire pour la finalité poursuivie par le traitement, traitement, en contrariété avec le principe de minimisation de la collecte imposé par le règlement européen. Cela risque de faire peser une charge trop importante sur les responsables de traitement et sous-traitants de données à caractère personnel, mais également de porter une atteinte injustifiée à la vie privée des personnes concernées. Enfin, un autre risque est de voir émerger des situations de conflits de lois inextricables entre le droit français et celui d'un autre État membre qui aurait choisi de retenir un autre critère pour l'application de sa loi nationale en complément du règlement européen.

lorsqu'elle sera appliquée en complément du règlement européen, sur des critères analogues à ceux prévus par ce dernier. Cette réécriture aura également pour effet d'uniformiser le champ d'application territorial de la loi de 1978 selon qu'elle est appliquée seule ou en complément du règlement, renforçant ainsi la lisibilité du texte. Quel est l'avis de la commission ? sollicite le retrait de cet amendement, qui vise à modifier le critère fixant le champ d'application territorial des règles françaises adaptant ou complétant le règlement. Voilà ! Au critère du lieu de résidence de la personne concernée par le traitement des données, il entend substituer plutôt le critère du lieu d'établissement du responsable de traitement. Ce changement est contraire à la position de la commission, qui a maintenu le critère de résidence. Comme le note justement l'étude d'impact du projet de loi, le « critère de l'établissement » aurait certes pour avantage premier de permettre au responsable de traitement de n'appliquer qu'un seul droit- cela permettrait de réduire certaines charges administratives et diminuerait la complexité juridique pour le responsable, et uniquement pour lui -, mais, dans une telle hypothèse, le droit applicable aux personnes concernées pourrait varier en fonction du lieu d'établissement principal du responsable de traitement ou de son sous-traitant. Concrètement, cela reviendrait à faire application du droit d'autres États membres pour des traitements de données qui touchent des résidents français. Je donne un exemple. Si l'Irlande choisit comme âge de consentement des mineurs, en ce qui concerne l'offre directe de services de la société de l'information, l'âge de treize ans, ou si elle exclut l'action de groupe pour la réparation des dommages, ces dispositions s'appliqueront aux résidents français pour l'utilisation de services tels que Google ou Facebook, dont le siège des filiales européennes se trouve en Irlande. Quel est

une innovation majeure par rapport à la directive de 1995. L'article 3 du règlement, comme cela vient d'être dit, prévoit en effet un double champ d'application. D'une part, ce règlement est applicable aux traitements effectués dans le cadre des activités d'un établissement par un responsable de traitement ou un sous-traitant dès lors que celui-ci se trouve sur le territoire de l'Union, peu importe que le traitement d'ailleurs ait lieu ou non dans l'Union. Il s'agit donc en quelque sorte d'un critère organique. D'autre part, le règlement est également applicable selon un critère matériel, peu importe que l'établissement soit alors sur le territoire de l'Union, dès lors que le traitement est effectué à l'égard des résidents européens. Il suffit alors que l'offre de biens ou de services à des personnes concernées se déroule dans l'Union ou que leur comportement dans l'Union soit suivi. Le règlement a donc une cohérence globale vis-à-vis des responsables de traitement présents dans ou en dehors de l'Union. Il précise à cet égard, à son considérant 14, qu'il devrait s'appliquer aux personnes physiques, indépendamment de leur nationalité ou de leur lieu de résidence en ce qui concerne le traitement de leurs données. Si son champ d'application est déjà défini par le RGPD,

en cas de divergences, compte tenu des choix différents dans l'exercice de ces marges de manoeuvre qui sont permises par le règlement. Les enjeux sont importants en termes de protection des droits fondamentaux des personnes concernées, mais également également d'attractivité des territoires, dès lors que la législation applicable peut constituer un critère très important pour une entreprise qui souhaite s'implanter à l'étranger. L'article 8 du projet de loi prévoit ainsi de retenir pour l'application des marges de manoeuvre, cela a déjà été dit, le critère de résidence de la personne concernée, à l'exception des traitements mentionnés à l'article 85.2 du règlement en matière de liberté d'expression et d'information, qui relèveraient du critère d'établissement du responsable de traitement. Son objet est donc clairement défini. L'amendement proposé, au contraire, laisse subsister, si vous me permettez cette expression, une forme d'oubli. En effet, le 1° du II tend à proposer un critère qui est centré sur la localisation, en France, du responsable du traitement. Le 2° traite du cas particulier du droit français qui s'applique en vertu du droit international public. Le 3° concerne enfin exclusivement le cas où le responsable de traitement n'est pas établi dans l'Union européenne. Or ce cas est déjà réglé à l'article 3.2 du RGPD. Ainsi, il manque, me semble-t-il, le plus important. Quel droit s'applique lorsque le responsable de traitement est dans l'Union européenne, mais hors de France, et que ses services s'appliquent à un résident en France Autrement dit, à quoi servent tous nos débats sur l'âge de consentement des mineurs ou sur les garanties relatives au NIR, aux données biométriques ou aux données de santé, si le droit qui est issu des marges de manoeuvre des autres États membres venait alors à s'appliquer en France directement

M. Jérôme Durain. Le règlement est applicable à partir du 25 mai 2018. L'ensemble des traitements existants devront donc être conformes au règlement à cette date. Le présent amendement a pour objet de prendre en compte la situation des traitements en cours dans une optique de sécurité juridique et de simplification, en particulier pour les acteurs économiques récents et de petite taille. Cet amendement s'inscrit dans l'esprit du considérant 171, qui prévoit déjà une série d'exceptions

l'avis du Gouvernement ?

Sur l'application dans le temps aux traitements en cours, le règlement a prévu uniquement le cas des accords conclus par les États membres. Lors des négociations, le gouvernement français avait voulu obtenir une clause relativement aux traitements en cours, sans succès. Le considérant 171 du règlement prévoit néanmoins que certains traitements qui sont mis en oeuvre conformément au droit national antérieur au 25 mai 2018 pourront bénéficier de la présomption de conformité au règlement jusqu'à leur modification, remplacement ou abrogation, à savoir, d'une part, les traitements ayant pour condition de licéité le consentement de la personne concernée si ce consentement a été donné dans les conditions prévues par le règlement et, d'autre part, les traitements soumis aux autorisations de la CNIL relatives à des transferts de données en dehors de l'Union européenne. Ainsi, le règlement ne permet pas une très grande souplesse si les traitements n'ont pas été modifiés au 25 mai 2018. Le projet de loi ne prévoit donc pas de mesure relative aux traitements en cours. La Commission européenne est d'ailleurs très vigilante sur ce point et pourrait sanctionner Toutefois, dans ses lignes directrices, le G29, le groupe de travail qui rassemble les « CNIL » européennes, donne une portée plus importante à ce considérant 171, puisqu'il estime qu'aucune analyse d'impact n'est nécessaire pour les opérations de traitement qui ont fait l'objet d'un examen par la CNIL. Par conséquent, il me semble que la question se réglera plutôt dans le cadre de la pratique de la CNIL. À cet égard, celle-ci a d'ores et déjà indiqué, par exemple, qu'une analyse d'impact ne sera pas exigée pour les traitements qui ont fait l'objet d'une formalité préalable auprès de la CNIL

Carrère. Cet amendement vise à renforcer les obligations de transparence des responsables de traitement et de leurs sous-traitants, afin d'améliorer l'information des personnes concernées par les traitements de données personnelles sur le droit applicable au responsable du traitement de ces données et à ses éventuels sous-traitants. Le maintien dans le règlement européen de marges de manoeuvre à la discrétion des États membres risque de laisser perdurer d'importantes différences en matière de protection des données personnelles au sein de l'Union européenne, ce qui pourrait induire le développement de pôles économiques dédiés à la sous-traitance des données personnelles

retrait de cet amendement, parce qu'il est en partie satisfait par l'article 13 du règlement général sur la protection des données, qui définit de façon exhaustive les obligations de transparence en faveur des personnes dont les données sont l'objet de traitement, notamment l'identité et les coordonnées du responsable du traitement et, le cas échéant, du représentant du responsable du traitement, les destinataires ou les catégories de destinataires des données. Cet amendement prévoit en outre des obligations supplémentaires qui ne sont pas du tout prévues par le RGPD et auxquelles je ne peux donc être favorable. Quel

chaque fois que cela est possible. En effet, le chiffrement de bout en bout, où seules les personnes autorisées à accéder aux données ont la clef, limite considérablement les risques d'intrusion.

dispose : « Le responsable du traitement est tenu de prendre toutes précautions utiles, au regard de la nature des données et des risques présentés par le traitement, pour préserver la sécurité des données et, notamment, empêcher qu'elles soient déformées, endommagées, ou que des tiers non autorisés y aient accès. » Notre amendement, à l'instar de celui qui vient d'être défendu par nos collègues du groupe LR, LR, tend à préciser la notion de « précautions utiles », en ajoutant que, chaque fois que cela est possible, les données devraient être chiffrées afin de n'être accessibles qu'au moyen d'une clef mise à la seule disposition des personnes autorisées à y accéder. Nous considérons en effet que le chiffrement des données de bout en bout est la seule technique à même de limiter les risques d'intrusion. Quel

peut également se révéler non pertinente pour certains traitements. En effet, le chiffrement ne constitue que l'une des mesures pour atténuer les risques inhérents au traitement afin de garantir la sécurité. L'article 32 du règlement prévoit ainsi que, « compte tenu de l'état des connaissances, des coûts de mise en oeuvre et de la nature, de la portée, du contexte et des finalités du traitement ainsi que des risques, [ ...], le responsable du traitement et le sous-traitant mettent en oeuvre les mesures techniques et organisationnelles appropriées afin de garantir un niveau de sécurité adapté aux risques, y compris entre autres, selon les besoins ». Parmi celles-ci figurent notamment la pseudonymisation et le chiffrement des données à caractère personnel. Il s'agit donc d'une mesure de sécurité parmi d'autres, qui ne saurait être imposée systématiquement au responsable de traitement. Il appartient à ce dernier, au regard du principe de responsabilisation, et sous le contrôle de la CNIL, d'apprécier laquelle de ces mesures est la plus appropriée à son traitement et au risque potentiel qu'il présente. Je mets aux voix l'amendement

Carrère. Vous connaissez tous les risques liés à la constitution de données sensibles à partir des données personnelles publiées volontairement pas des usagers d'outils numériques et de réseaux sociaux. Il peut ainsi exister des profilages à partir de « réactions » ou de commentaires laissés sur tel ou tel article, telle ou telle page internet, qui peuvent permettre d'établir des bases de données comportant des indications sur les orientations sexuelles d'une personne ou ses convictions politiques. D'une part, ces profilages peuvent se révéler de simples extrapolations algorithmiques et, d'autre part, en agissant de la sorte, les utilisateurs n'ont pas nécessairement la volonté de rendre publiques les données concernées. Il apparaît que ce risque est insuffisamment pris en compte, tant dans le droit interne qu'en droit européen. C'est pourquoi nous proposons d'introduire cette modification. cet amendement, qui tend à donner au législateur la possibilité d'interdire le traitement de données sensibles rendues publiques. Outre qu'il ne précise pas lui-même les cas où une telle interdiction devrait s'appliquer, semble fusionner les régimes applicables à deux types différents de données : d'une part, le régime applicable aux données personnelles, pour lesquelles la personne a consenti au traitement- ces données peuvent ne pas avoir été rendues publiques le régime applicable aux données personnelles qui sont « manifestement rendues publiques » par la personne concernée- elles peuvent l'être sans un consentement exprès et verbalisé de la personne au sens du règlement général sur la protection des données. De plus, le présent amendement introduirait une restriction qui ne figure pas dans le règlement ; je vous propose de nous en tenir à la formulation de celui-ci.

de préserver la confiance des citoyens dans la justice et d'assurer aux justiciables une sécurité juridique. Malheureusement, aujourd'hui encore, le conservatisme s'oppose au mouvement de consécration de de la transparence de notre système judiciaire, notre commission ayant adopté un amendement visant à anonymiser les noms des magistrats et des avocats. Pourtant, le Conseil national des barreaux s'est opposé à l'unanimité à l'anonymisation des avocats dans les jugements dans une résolution du 3 février 2017. Dans le même sens, M. Louvel, premier président de la Cour de cassation, et les premiers présidents des cours d'appel se sont prononcés contre cette mesure. La CNIL s'est également prononcée contre la mesure dès 2001, et son avis est suivi dans toute l'Union européenne. Plus récemment, le rapport du professeur Loïc Cadiet, rendu en mai 2017, a considéré dans son point n° 71 que « l'occultation du nom du nom du magistrat reviendrait à cacher un des principaux acteurs du fonctionnement de l'institution judiciaire et ne garantirait plus la fiabilité et l'intégrité des données ouvertes- -, ce qui constitue alors un obstacle aux objectifs poursuivis par la loi ». L'anonymisation va contre le sens de l'histoire, mes chers collègues. Nous souhaitons donc revenir à la rédaction initiale du texte. est défavorable, car cet amendement vise à revenir intégralement au texte du projet de loi initial en supprimant tous les apports de la commission. L'objet de l'amendement ne mentionne que les dispositions votées concernant des décisions de justice. C'est oublier que l'article 11 ne concerne pas seulement ce sujet, mais également le régime général de licéité des traitements de données pénales et, plus particulièrement, la liste des personnes, y compris morales de droit privé, autorisées à mettre en oeuvre des fichiers concernant les infractions ou les condamnations pénales. Cet article adopté par la commission vise par exemple à permettre de maintenir le régime d'autorisation préalable des fichiers en matière pénale. Il convient donc de conserver les apports de la commission des lois.

contrairement à ce que l'objet de l'amendement laisse suggérer, le rapport Cadiet n'a pas pris position en faveur du maintien du nom des magistrats ; il a examiné les arguments pour et les arguments contre. Selon ce rapport, « la mention des noms des magistrats dans les décisions diffusées en mettrait à mal les principes » d'indépendance et de procès équitable. Le rapport concluait : « En définitive, il semble que les seules personnes qui, en dehors des parties et des juridictions, pourraient avoir un intérêt réel à connaître les noms des juges, seraient celles qui souhaiteraient porter à leur encontre des critiques personnelles, souvent malveillantes et injustifiées, voire discriminatoires, ou même s'en prendre à leur sécurité physique. « En effet, outre qu'elle ne présente aucune plus-value, la diffusion des noms des magistrats exposerait la justice et les juges à plusieurs risques principaux. » Il y a en effet un risque de, c'est-à-dire de stratégies délibérées des justiciables pour obtenir un juge en particulier, mais également un risque que les magistrats soient pris pour cibles, qu'il existe des tentatives de déstabilisation contre eux, voire d'atteinte à leur sécurité. « En somme, loin d'aboutir à favoriser la confiance du justiciable dans la justice, l'indication des noms des magistrats conduirait à l'affaiblir, sans concourir aux objectifs poursuivis par l'» Nous Nous ne parlons ici que des magistrats, mais les policiers et les greffiers qui interviennent au cours de la procédure et sont mentionnés dans le jugement doivent également, avec un fichier en facilement réutilisable, faire l'objet d'un procédé visant à prévenir tout risque de réidentification des personnes concernées.

Par cet amendement, le Gouvernement souhaite rétablir, pour l'essentiel, l'article 11 tel qu'il est issu des débats à l'Assemblée nationale. La rédaction retenue par la commission des lois ne nous semble en effet pas satisfaisante, car elle retient une définition des données d'infraction différente de celle de l'article 10 du RGPD, qui est impérative. En outre, il est nécessaire de revenir à la rédaction adoptée par l'Assemblée nationale s'agissant des personnes morales de droit privé collaborant au service public de la justice. En effet, la commission des lois a ajouté une condition leur permettant de traiter des données d'infraction, à savoir que leurs missions doivent avoir été confiées par la loi. Si je comprends la démarche de la commission, qui souhaite renforcer la protection de ce type de données, pour autant, la rédaction retenue est trop restrictive. Elle exclurait ainsi les associations d'aide aux victimes, qui bénéficient d'un agrément du ministère de la justice sans que des dispositions législatives consacrent leur mission. Par ailleurs, le présent amendement supprime le renvoi à un décret en Conseil d'État pris après avis de la CNIL pour définir les modalités selon lesquelles les personnes physiques ou morales peuvent traiter des données d'infraction pour leur permettre de préparer et, le cas échéant, d'exercer et de suivre une action en justice. Dans sa décision du 29 juillet 2004, le Conseil constitutionnel a précisé que les garanties appropriées et spécifiques doivent être fixées dans la loi. Les garanties qui figurent dans le présent projet de loi en termes de durée de conservation et de proportionnalité de la finalité suffisent à répondre aux conditions fixées par le Conseil constitutionnel, sans qu'il soit besoin de définir des durées maximales de conservation des informations enregistrées, les catégories de personnes autorisées à être destinataires de tels traitements ou encore les conditions de cette de cette transmission. Le Conseil d'État a d'ailleurs estimé que les précisions apportées par le projet de loi n'appelaient pas de réserve. Enfin, le présent amendement supprime le régime d'autorisation préalable par la CNIL avec une possibilité de décision unique, qui avait été réintroduit par la commission des lois. Un tel régime va en effet à l'encontre de l'objectif de non-surtransposition souhaité par le Gouvernement et de la philosophie du règlement européen, qui vise à alléger les formalités préalables. Cet allégement va de pair, en contrepartie, avec un accroissement du pouvoir de sanction de la CNIL. L'équilibre auquel était parvenue l'Assemblée nationale sur cette disposition doit être maintenu.

est très défavorable. Cet amendement vise d'abord à étendre considérablement, sans aucune forme de garantie, la liste des personnes pouvant mettre en oeuvre des traitements d'infractions pénales, de condamnations ou de mesures de sûreté dès lors qu'ils s'effectuent « sous le contrôle de l'autorité publique », sans autre précision. Cela s'entend hors des fichiers directement mis en oeuvre par les autorités publiques qui, eux, restent mentionnés au 1° de l'article 9 de la loi de 1978. Avec la suppression de l'ensemble du régime d'autorisation préalable des fichiers prévu actuellement par l'article 25 de la loi du 6 janvier 1978, le projet de loi tend désormais à encadrer les fichiers mis en oeuvre par l'État plus strictement que les fichiers mis en oeuvre par des personnes physiques ou morales. C'est paradoxal ! en matière pénale, les risques pour les personnes, notamment d'atteinte à la vie privée et de négation du droit à l'oubli, peuvent provenir de l'utilisation à des fins privées de telles données.

Je rappelle que, selon le considérant 19 du règlement, « les États membres devraient pouvoir maintenir ou introduire des dispositions plus spécifiques » quand il s'agit de maintenir un niveau élevé d'exigences en matière de protection des données personnelles. Le règlement n'impose aucunement de baisser notre niveau d'exigence. Ce n'est pas de la surtransposition quand il s'agit de maintenir nos règles actuelles ! S'agissant de la directive, le considérant 15 prévoit ainsi Le rapprochement des législations des États membres ne devrait pas conduire à un affaiblissement de la protection des données à caractère personnel qu'elles offrent mais devrait, au contraire, avoir pour objectif de garantir un niveau élevé de protection dans l'Union. Il convient que les États membres ne soient pas empêchés de prévoir des garanties plus étendues que celles établies dans la présente directive pour la protection des droits et des libertés des personnes concernées à l'égard du traitement des données à caractère personnel par les autorités compétentes. Cet amendement vise enfin à supprimer toutes les garanties introduites par la commission s'agissant des fichiers en matière pénale mis en oeuvre par toute personne physique ou morale. Ces garanties n'empêcheraient pas les associations de victimes de tenir de tels fichiers, puisque leurs missions légales sont fixées par la loi, notamment par l'article 10-2 du code de procédure pénale. Les garanties prévues par la commission constituent, selon moi, le strict minimum pour répondre aux exigences constitutionnelles et, notamment, à sa décision n° 2004-499 DC du 29 juillet 2004. Il est indispensable que le décret prévoie la durée maximale de conservation des informations enregistrées et que soient précisées les catégories de personnes, par exemple les associations de victimes, autorisées à être destinataires de tels traitements. Je rappelle que, en 2004, le Conseil constitutionnel avait censuré une disposition similaire en raison de l'absence de précision sur les limites susceptibles d'être assignées à la conservation des mentions relatives aux condamnations. L'élargissement de la possibilité de mettre en oeuvre de tels traitements par les personnes morales, et à l'époque avec des formalités préalables, avait été censuré par le Conseil, qui avait considéré que, en raison de l'ampleur que pouvait revêtir les traitements de données personnelles ainsi mises en oeuvre et de la nature des informations traitées, une telle disposition pourrait affecter, par ses conséquences, le droit au respect de la vie privée et les garanties fondamentales accordées aux citoyens pour l'exercice des libertés publiques. La rédaction de cette disposition est imprécise, reste muette sur les conditions dans lesquelles les données traitées pourraient être partagées ou cédées, ou encore si pourraient y figurer des personnes sur lesquelles pèse la simple crainte qu'elles soient capables de commettre une infraction. Rien n'est dit sur les limites susceptibles d'être assignées à la conservation des mentions relatives aux condamnations.

La rédaction proposée par la commission des lois impose que la diffusion des décisions de justice prévienne tout risque de réidentification. Il s'agit là d'un objectif impossible à atteindre, sauf à effacer des parties entières des décisions de justice

rappelle que la prévention absolue de la réidentification est impossible en pratique, car les décisions de justice sont des documents très construits, qui contiennent de nombreuses données réidentifiantes.

et non de résultat. Cette analyse est approuvée par la CNIL et par les cours suprêmes, qui ont concouru à cette mission. Il faut donc aller, me semble-t-il, vers une protection adaptée de la vie privée des personnes concernées par les décisions Les mentions d'identification contenues dans les décisions doivent être supprimées et la réidentification doit être, bien entendu, difficile à effectuer.

est défavorable. Si la commission a modifié le régime de l'des décisions de justice, c'est tout simplement parce que les magistrats ont très largement demandé des règles protectrices en matière d'anonymisation des décisions, pour que l'on ne puisse pas dresser et diffuser des profils de juges. Nous avons tout de même le devoir de protéger les professionnels de la justice : c'est un minimum, me semble-t-il. Le rapport Cadiet est très clair quant au risque que l'on prend en publiant le nom des magistrats en. En somme, loin d'aboutir à favoriser la confiance du justiciable dans la justice, l'indication des noms des magistrats conduirait à l'affaiblir, sans contribuer aux objectifs visés à travers l'. L'USM, qui représente plus de 70 % des magistrats, l'a très clairement réaffirmé : la non-anonymisation des décisions de justice et la prévention du risque de non-réidentification des magistrats devaient être des garanties inscrites dans la loi. Dès lors, une telle disposition ne peut passer simplement par un décret. Pourquoi effacer également le nom des avocats ? Lors des travaux de la mission d'information sur le redressement de la justice, certains se sont émus des risques de individuel des avocats, en fonction de leur taux de réussite dans les dossiers qu'ils plaident, sans considération, évidemment, ni pour la nature de l'affaire ni pour sa difficulté. J'y insiste, ces dispositions ne remettent pas du tout en cause le principe de publicité des jugements, mais définissent les modalités de leur mise à disposition massive en, compte tenu des utilisations qui pourraient en être faites grâce aux nouvelles technologies.

Elles comportent les noms des magistrats, des avocats et des parties. Il ne s'agit pas ici de décider si l'on doit les rendre publiques ou pas : elles sont publiques, et elles le resteront. Il s'agit ici de décider quelle extension nous devons donner à la mise à disposition, en masse, des décisions de justice. L'des décisions de justice a été décidée. Nous nous sommes prononcés sur cette question. Le premier président de la Cour de cassation anime un travail très important pour permettre la mise en oeuvre de cet, et il faut lui en rendre hommage. Cela étant, il faut aussi avoir à l'esprit les implications d'une exploitation à grande échelle, par des algorithmes, d'un certain nombre de données qui permettraient de déterminer à l'avance où l'on a le plus de chance d'obtenir satisfaction,

de la justice, dans l'intérêt des justiciables, dans l'intérêt aussi des auxiliaires de justice, sans pour autant permettre, à grande échelle,

Mme la ministre.

Ce que nous proposons, c'est de rétablir la rédaction adoptée par l'Assemblée nationale, en vertu de laquelle les traitements mis en oeuvre ne doivent avoir ni pour objet ni pour effet de permettre la réidentification des personnes concernées.

condition nécessaire pour leur permettre d'exercer utilement leur activité d'étude et d'analyse du droit. Ces acteurs ne sauraient être assimilés aux réutilisateurs entendus dans leur acception la plus large. Ils doivent pouvoir disposer d'un accès distinct aux informations publiques figurant dans les jugements mentionnés à l'article L. 10 du code de justice administrative et dans les décisions mentionnées à l'article L. 111-13 du code de l'organisation judiciaire.

Cette rédaction impose certaines conditions spécifiques aux traitements autres que ceux qui sont menés à des fins archivistiques, historiques, scientifiques et statistiques. Or ces traitements sont déjà soumis au régime de droit commun prévu par le RGPD. Quel est l'avis de la commission ? Avis favorable.